Gabriel Attal, que j'ai l'honneur et le plaisir de remplacer aujourd'hui pour l'examen en nouvelle lecture de ce projet de loi de règlement de l'année 2021. S'agissant de ce texte, beaucoup de choses ont été dites lors de l'examen en première lecture. Permettez-moi néanmoins d'y revenir brièvement. À la faveur de l'amélioration de la situation sanitaire, l'année 2021 a été celle de la sortie progressive du « quoi qu'il en coûte », de la reprise économique et du début du redressement de nos comptes. encore été marquée par de très fortes turbulences sur les plans sanitaire et économique. Cette instabilité explique d'ailleurs le montant des reports de crédits effectués l'année dernière, soit 24,6 milliards d'euros, sur lesquels nous avons eu l'occasion de nous expliquer lors de la première lecture. 2021 a aussi été l'an un du redressement des comptes. Sous la conduite de Bruno Le Maire et d'Olivier Dussopt, notre déficit public a diminué de 2,5 points de PIB, passant de 8,9 % à 6,4 %. Pour autant, cette sortie progressive du « quoi qu'il en coûte » n'a jamais été conduite au détriment des Français, que nous avons le devoir impérieux de protéger des aléas économiques. Durant cette période, nous avons tout fait pour ne pas ajouter la vulnérabilité financière à la vulnérabilité sanitaire. S'agissant de la protection des ménages, je veux mentionner les 3,8 milliards d'euros mobilisés pour verser une indemnité inflation de 100 euros à 38 millions de foyers, ou encore les 600 millions d'euros engagés pour verser un chèque énergie exceptionnel à 5,6 millions de foyers de foyers modestes juste avant les fêtes de fin d'année. Cependant, on ne protège pas les individus sans aider les entreprises qui les emploient. Nous avons donc, durant ces mois de pandémique, constamment adapté nos dispositifs. Je pense en particulier à l'activité partielle, dont ont bénéficié 3,5 millions de salariés. Globalement, nous avons mobilisé plus de 34 milliards d'euros dans le cadre de la mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire ». Ce faisant, nous n'avons pas fait de cadeaux aux entreprises, comme j'ai pu l'entendre : nous leur avons permis de tenir le choc, de ne pas manquer de trésorerie, de continuer d'investir et d'embaucher.

et fort pour accélérer la transition énergétique, pour renforcer la compétitivité et le dynamisme de nos industries, mais aussi pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Assumer la fin du « quoi qu'il en coûte » sans laisser les agents économiques à la merci de la crise : voilà la ligne de crête sur laquelle le Gouvernement avance. Et je crois pouvoir le dire, cette politique a fait la preuve de son efficacité l'année dernière. En faisant le choix de la protection et de la relance, nous avons fait le choix de la croissance et de l'emploi. Avec une croissance de 6,8 % l'année dernière, notre pays fait 1,4 point de mieux que la moyenne de la zone euro. Certains ont voulu y voir uniquement un effet de rattrapage, sans jamais concéder le moindre satisfecit s'agissant de notre gestion. Je veux simplement dire que nous pourrions de temps en temps nous réjouir lorsque notre pays réussit, car c'est le fruit du travail de tous. S'agissant de la situation de l'emploi, celle-ci n'a jamais été si favorable depuis 2008, avec un taux de chômage ramené à 7,3 % de la population active et un chômage des jeunes au plus bas depuis quarante ans. Là aussi, réjouissons-nous que notre pays aille mieux, après des décennies de chômage de masse. Grâce à la vigueur de la reprise, nous avons pu compter sur un surplus de recettes fiscales. Par rapport à la loi de finances initiale, ce sont 37,9 milliards d'euros supplémentaires que nous avons encaissés, grâce au dynamisme de l'impôt sur les sociétés, de la TVA et de l'impôt sur le revenu. À l'occasion de la première lecture, certains d'entre vous ont cherché à démontrer que ce surplus était uniquement lié aux circonstances et à l'effet de l'inflation, sans jamais admettre que notre politique de compétitivité et d'attractivité avait contribué, sans doute, à la bonne santé de nos entreprises et donc au rendement de l'impôt sur les sociétés, et ce malgré une baisse de son taux. Là aussi, j'aurais aimé que nous puissions nous retrouver sur ce constat. Finalement, et en dépit des critiques formulées, l'année 2021 aura donc été celle de la validation de la stratégie du Gouvernement : soutenir l'activité économique et faire diminuer le chômage, pour plus de croissance et plus de rentrées fiscales. La parole

2019. D'ailleurs, nos performances ont été moins bonnes que celles de nos partenaires européens. Rétrospectivement, on peut observer qu'en 2021 nous avons subi un certain nombre de chocs économiques,

En tout état de cause, ce rattrapage économique a eu un coût, monsieur le ministre, celui de la dégradation de nos comptes publics. Les recettes publiques ont en effet été sous-évaluées lors de l'examen du PLFR de fin de gestion en 2021,

d'euros, s'accordant là un brevet de bonne conduite pour sa gestion. Par ailleurs, si les dépenses publiques sont inférieures de 10 milliards d'euros à la prévision retenue dans le PLFR de fin de gestion, leur montant nous éloigne encore très fortement des objectifs inscrits en loi de programmation des finances publiques, et notre déficit est aujourd'hui principalement supporté par l'État, tandis que les collectivités locales parviennent quasiment à l'équilibre et que les administrations de sécurité sociale ont divisé par plus de deux leur déficit.

supérieur à 170 milliards d'euros, parce que nous subissons toujours une augmentation de nos dépenses : 420 milliards d'euros pour moins de 250 milliards d'euros de recettes.

Or je n'ai pas le sentiment que cela soit perçu comme une situation exceptionnelle, puisqu'aucune diminution de dépenses n'est à ce jour prévue. Du point de vue budgétaire, le montant extraordinaire des reports de crédits opérés en 2021 est très contestable : plus de 36 milliards d'euros,

Pour toutes ces raisons, et par cohérence avec le vote du Sénat en première lecture, je propose que le Sénat n'adopte pas le projet de loi de règlement et d'approbation des comptes de l'année 2021.

En revanche, nous ne voterons pas le présent projet de loi de règlement, car il traduit une dérive des finances publiques marquée par une forte augmentation du déficit structurel. Celui-ci aura en effet doublé sur la durée du quinquennat, passant de 72 milliards d'euros à 145 milliards d'euros ! Malgré un fort rebond des recettes fiscales, le déficit de l'État est, en 2021, quasiment identique à son niveau de 2020, année dont chacun mesure le caractère exceptionnel. Nous regrettons que le Gouvernement n'ait pas utilisé ces recettes supplémentaires pour réduire l'endettement, comme l'y invitait la commission des finances du Sénat. Notre dette publique approche désormais les 3 000 milliards d'euros. Elle s'est accrue de 665 milliards d'euros en cinq ans, et le PLFR, malheureusement, ne fera qu'aggraver la situation. La cote d'alerte, pour reprendre une expression de notre ministre de l'économie et des finances, était donc atteinte bien avant cette année. Cette incapacité à maîtriser nos finances publiques est d'autant plus inquiétante que nous assistons désormais à une remontée des taux d'intérêt. Les taux à dix ans, qui sont restés négatifs et pratiquement constants depuis 2019, sont devenus positifs. À la mi-juin, ils étaient proches de 2 % et pourraient atteindre 3 % à la fin de décembre. Nous le voyons avec le collectif budgétaire que nous sommes en train d'examiner en parallèle, la seule charge de la dette s'est déjà alourdie de 15 milliards d'euros en 2022 Nous ne pouvons plus continuer à vivre dans un tel déni de réalité. Nous ne pouvons plus, vous ne pouvez plus, monsieur le ministre, vous abriter éternellement derrière la crise sanitaire et son caractère exceptionnel. Le dérapage de nos finances publiques n'est pas imputable à la seule crise de la covid-19. Les dépenses courantes, indépendantes de la crise sanitaire et du plan de relance, ont augmenté en 2021 de 17,6 milliards d'euros, le tout sans la moindre économie en regard. Le rapport de la Cour des comptes est, à cet égard, cinglant et éloquent quant au manque d'ambition réformatrice du Gouvernement. Les quelques mesures du début de quinquennat n'auront pas permis au pays d'affronter la crise covid et, désormais, l'inflation, dans de bonnes dispositions financières. Nous regrettons que, dans le même temps, l'État n'ait pas répondu aux difficultés financières des collectivités locales. Je rappelle qu'elles ont subi près de 7 milliards d'euros de pertes en 2020 et 2021, dont 3,2 milliards d'euros pour les seules communes et leurs groupements, du fait de la covid. Les réponses apportées par le Gouvernement ont été, sur ce point, clairement insuffisantes, malgré les demandes du Sénat. En dépit des dénégations du Gouvernement, les faits sont là : la Cour des comptes indique que, à la fin de 2021, plus de 45 % des communes disposent d'un niveau d'épargne qui reste inférieur à celui de 2019. Le refus initial du Gouvernement de prévoir dans le cadre du projet de loi de finances rectificative que nous examinons actuellement une compensation pour la revalorisation du point d'indice et des dépenses énergétiques démontre une nouvelle fois le peu d'attention que celui-ci porte à nos collectivités. D'autres raisons justifient notre position d'abstention. Elles tiennent notamment aux conditions d'examen du texte, qui ne permettent pas au Parlement de remplir convenablement sa mission d'évaluation et de contrôle. Premier texte financier du second quinquennat, le projet de loi de règlement est examiné à la hâte, puisque le texte a été déposé le 4 juillet, alors qu'il aurait dû l'être avant le 1 juin, en application de l'article 46 de la LOLF. On est loin des bonnes intentions proclamées à l'attention du Parlement, et notamment du Sénat, par le Gouvernement. Cette situation n'est pas admissible, à plus forte raison quand on connaît l'état de nos comptes publics. Une loi de règlement est vidée de son utilité lorsque le Parlement ne dispose pas du temps nécessaire pour exercer ses prérogatives de contrôle et d'évaluation. Au-delà de ces problèmes de calendrier, il n'est pas admissible non plus que soient à ce point malmenés les principes budgétaires et, à travers eux, la portée de l'autorisation parlementaire. Qu'il y ait plus de 20 milliards d'euros de crédits reportés et des crédits ayant servi à financer d'autres programmes budgétaires que ceux prévus par la représentation nationale illustre, une fois de plus, le manque de respect du Gouvernement pour le Parlement.

nous voici de nouveau réunis pour examiner les montants définitifs des recettes et dépenses du budget de l'État en 2021. Il s'agit d'un passage obligé, un exercice de constatation pour l'essentiel, mais qui nous permet de dresser un bilan financier de l'année précédente précédente et, au passage, d'observer les écarts entre les résultats et les prévisions de la loi de finances initiale. Et des écarts, il y en a eu ... Secouée par une crise sanitaire dont nous avions vainement espéré l'achèvement dès 2020, la France a subi encore 2021 les remous puissants de la pandémie et de la crise économique qui a suivi. Notre croissance a également connu un rebond historique cette année-là, atteignant 7 % du PIB et établissant un record depuis une cinquantaine d'années, après la récession tout aussi historique de 2020. Malgré cette croissance, le déficit budgétaire de l'État atteint le niveau abyssal de 170,7 milliards d'euros, ce que ne suffit pas à rattraper le bon niveau des recettes fiscales net, qui ont retrouvé dès 2021 leur niveau d'avant-crise. Les dépenses brutes subissent une hausse de plus de 16 milliards d'euros, portant le total à 557 milliards d'euros pour 2021, principalement sur les postes de dépenses « Enseignement scolaire », « Défense », « Engagements financiers de l'État » et, bien sûr, le « Plan d'urgence face à la crise sanitaire ». Les objectifs définis en 2017 en loi de programmation des finances publiques prévoyaient pour 2021 un déficit effectif de 0,9 % du PIB. Les mesures exceptionnelles activées au printemps 2020 ont naturellement bouleversé la donne, aboutissant à un déficit de 6,4 %, très loin de l'objectif fixé quatre ans plus tôt. Ce n'est pas du tout la trajectoire qu'avait envisagée le Gouvernement, pas plus que le Parlement. L'ambition d'un redressement rapide des finances publiques s'est éloignée, mais, dans des circonstances aussi exceptionnelles, il était indispensable de lever certains verrous, sous peine de voir notre économie s'effondrer durablement. Le « quoi qu'il en coûte » a donc coûté très cher au budget de la France, mais a permis d'épargner à notre économie des stigmates durables, dont elle ne se serait pas remise. Par ailleurs, si l'incertitude a dominé les orientations budgétaires de 2021, force est de constater que la guerre en Ukraine et la crise de l'énergie ne nous permettront pas de prévoir avec plus de garanties les finances de l'État pour 2023. alors que nous venons d'adopter le projet de loi sur le pouvoir d'achat, qui prévoit plus de 20 milliards d'euros de dépenses supplémentaires en 2022, bientôt complété par le projet de loi de finances rectificative, préoccupations demeurent pour notre groupe : le retour à des finances plus saines, et, bien sûr, le soutien financier aux collectivités territoriales, avec, toujours en ligne de mire, l'indispensable investissement pour un avenir plus durable pour notre pays.

Ce texte, qui traduit l'exécution budgétaire de l'exercice passé, n'ayant pas connu d'évolution depuis le 19 juillet dernier- on voit assez mal comment il aurait pu en être ainsi -, appellera de notre part une conclusion identique. Je ne reviens pas sur les circonstances de son dépôt tardif. Nous avons tous pu largement nous exprimer à ce sujet, et j'ai bien noté l'engagement du ministre des comptes publics à respecter à l'avenir les dates prévues par la LOLF. Si je peux donner quitus sur ce point, j'ai été moins convaincue par le reste des arguments sur le fond. Certes, la crise sanitaire a bouleversé considérablement notre fonctionnement habituel certes, des dispositifs exceptionnels ont été mis en oeuvre pour soutenir notre économie, et le « quoi qu'il en coûte » était nécessaire, mais la crise n'explique pas tout. tout. J'ai bien noté, monsieur le ministre, les explications du Gouvernement concernant la dégradation du solde structurel. Si l'on peut tout à fait entendre la part prise par les dispositions de soutien d'urgence, qui n'est pas contestable, il est impossible de ne pas s'interroger sur votre obstination à refuser toute nouvelle recette fiscale. Ce solde témoigne donc bien de l'impasse fiscale de ce gouvernement, qui refuse de faire contribuer les entreprises et les plus aisés à la solidarité nationale, alors même que, rapport après rapport, l'ensemble des analyses démontrent l'inefficacité de la théorie du ruissellement, pourtant encore mise en avant aujourd'hui. Et ce ne sont pas les propos tenus par le ministre de l'économie et des finances lors des discussions générales du projet de loi sur le pouvoir d'achat et du PLFR qui risquent de nous rassurer sur ce point. Alors que vous évoquez une stratégie vertueuse pour nos finances publiques, j'ai la faiblesse de croire que les 50 milliards d'euros d'impôt auxquels le Gouvernement a renoncé ces dernières années auraient été fort utiles à l'heure où, toujours selon le ministre de l'économie et des finances, « nous avons atteint la cote d'alerte sur les finances publiques ». Non, monsieur le ministre, cette stratégie n'est pas vertueuse pour nos finances ; elle n'est pas non plus redistributive pour nos concitoyens. de loi de règlement illustre bien une politique de l'offre centrée sur les plus aisés, oubliant sur le bord de la route les plus fragiles d'entre nous. Une politique de la demande eût été possible : il aurait fallu pour cela prendre conscience de l'urgence sociale de notre pays et oublier les cadeaux fiscaux généreusement octroyés depuis 2017. On parle souvent de l'ISF comme d'un symbole, mais un symbole à 5 milliards d'euros mérite que l'on s'y intéresse ! La Cour des comptes a par ailleurs pointé dans son rapport le montant très élevé des niches fiscales- plus de 90 milliards d'euros en 2021. Peut-être y aurait-il, là aussi, quelques pistes intéressantes. Nous aurons, j'en suis certaine, l'occasion d'en rediscuter dans les mois qui viennent. Puisque nous en sommes aujourd'hui à l'exécution des comptes 2021, la Cour n'a pas non plus manqué de relever les entorses aux principes d'annualité et de spécialité budgétaires, qui affaiblissent considérablement la portée de l'autorisation parlementaire. En effet, le niveau de report de crédits, la confusion entre les exercices budgétaires, l'utilisation répétée de crédits de programmes budgétaires pour financer des dépenses relevant d'autres programmes nuisent grandement à la lisibilité de ce texte. Ce manque de sérieux et de clarté sert, il est vrai habilement, à masquer les échecs d'une politique gouvernementale très éloignée de la satisfaction affichée par l'exécutif.

Il me semble pourtant que l'objectif annuel était de 800 000 logements. Nous le voyons bien, il y a loin de la coupe aux lèvres, surtout que la Cour, encore elle, indique que seuls 2 500 logements étaient sortis de la catégorie « passoire thermique » en 2021 grâce à ce dispositif. Ce dernier exemple illustre bien la méthode employée dans la présentation de ces comptes 2021. Ce projet de loi de règlement n'est pas seulement une exécution budgétaire ; il va bien au-delà. Il est la traduction d'une méthode qui remet en cause la mission de contrôle du Parlement, mais aussi, et surtout, il signe l'entêtement idéologique du Gouvernement dans une politique purement libérale, pourtant mise à mal et sans résultat. Comme en première lecture, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera contre ce projet de loi de règlement et d'approbation des comptes de 2021. La parole

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'année qui vient de s'écouler n'était comparable à aucune autre ; c'est pourquoi le budget qui l'accompagnait a été nécessairement exceptionnel. Malgré ce contexte, le projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2021 vient entériner la politique résolument réaliste du Gouvernement. Réaliste, notre politique l'était quand nous avons répondu à l'urgence sociale qui résultait de la crise sanitaire, alors que nous ne pouvions détourner le regard

concitoyens sans agir. Le « quoi qu'il en coûte » a eu un prix, mais ce qu'il a permis de sauver n'en avait pas. Je mets au défi quiconque de nier l'importance du rôle qu'ont joué les mesures du Gouvernement pour protéger le pouvoir d'achat des Français lors de la crise sanitaire.

Incertitudes, doutes et imprévisions caractérisaient la situation économique et financière de notre pays : le Gouvernement y a répondu avec fermeté, volonté et sincérité. La longue période durant laquelle nous avons su protéger les Français ainsi que notre économie ne doit cependant pas nous faire perdre de vue notre ligne politique et nos engagements : une action publique efficace et responsable, finançable et Nous devons maintenant remettre nos comptes en ordre en retrouvant un déficit inférieur à 3 % d'ici à 2027 afin de mettre en place un projet politique responsable et de transmettre une situation financière pérenne aux générations futures. La réduction de ce déficit est possible par notre politique d'emploi et de croissance qui, en plus de permettre un assainissement de nos comptes, est la seule solution pour améliorer le pouvoir d'achat des Français. Cette politique n'est pas seulement une vue de l'esprit ou idéologique : elle s'incarne positivement dans notre pays, puisque notre taux de chômage est au plus bas depuis 2008.

des recettes fiscales a permis une baisse du déficit public de plus de 2 %. Nous pouvons faire l'objet de critiques, positives comme négatives, c'est l'essence même de notre démocratie ; chacun comprend bien pourtant que nous avons agi au mieux, contraints par une situation économique et sanitaire dans laquelle nous avons su à la fois éviter la misère tant redoutée et relancer la croissance tant convoitée. En définitive, ce projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes 2021 ne constitue pas une approbation totale de chacune des dépenses effectuées l'année passée, mais plutôt la ratification d'une gestion de crise nous permettant d'éviter collectivement la catastrophe économique et sociale. C'est pourquoi le groupe RDPI le votera. La parole est à M. Jean-Pierre

nous examinons depuis hier le projet de loi de finances rectificative pour l'année en cours, nous débattrons demain des grandes orientations budgétaires pour le quinquennat qui s'ouvre et, cet après-midi, nous discutons donc du projet de loi de règlement des comptes pour l'année précédente.

Pour renforcer le travail entre le Gouvernement et le Sénat, nous attendrons donc le prochain texte budgétaire ; espérons que cela soit possible dès le de ce projet de loi de règlement, le désaccord en CMP ne change rien : contester la facture après qu'elle a été réglée ne rend pas plus riche. En l'espèce, la facture a été salée. Le déficit s'est établi en 2021 à 6,4 % du PIB, notre dette publique, qui représente 113 % du PIB, atteint un niveau inquiétant, bien plus près des 120 % que des 60 % prévus par nos engagements européens. Cela aurait pu être encore pire si nous n'avions pas eu quelques bonnes nouvelles : le dynamisme de la croissance, finalement estimée à près de 7 % du PIB, et le recul du chômage ont significativement augmenté les recettes publiques. Nous pouvons nous en réjouir.

il est important de le rappeler, car, à trop noircir le tableau, on risque de regretter le soutien total de l'État à l'économie, aux entreprises et aux salariés. Or cela ne serait pas la meilleure façon de préparer l'avenir. Il faut le dire et le rappeler : la France a bien géré la crise les mesures que nous avons collectivement décidé de mettre en oeuvre ont permis de protéger les salariés et les entreprises dans une crise sans précédent. Les Français comptaient sur l'État et celui-ci a été au rendez-vous. Alors que les tensions sociales resurgissent de toutes parts, nous avons su préserver le pacte républicain. Il faudra désormais se mettre à l'oeuvre, travailler plus et gagner plus, pour ne pas laisser les prochaines générations payer l'addition du « quoi qu'il en coûte Nous devons tourner cette page, mais nous pouvons nous réjouir de l'avoir écrite collectivement. En tout état de cause, le groupe Les Indépendants-République et Territoires votera majoritairement en faveur de ce projet de loi de règlement, comme il l'avait fait en première lecture.

étayés par des auditions, lors de la discussion du projet de loi de finances.

Le déficit budgétaire reste très élevé et vous reportez des crédits non consommés, à hauteur de 23 milliards d'euros, de 2021 vers 2022, ainsi que l'a noté la Cour des comptes. Vous dérogez ainsi au principe de l'annualité budgétaire. Peut-être constituez-vous une cagnotte

9,2 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté dans notre pays, et la crise du covid a créé de nouveaux vulnérables, comme l'indique la Fondation Abbé Pierre. Les mesures de soutien à l'activité ont protégé les salariés, mais essentiellement ceux qui bénéficiaient d'un emploi stable et beaucoup moins les populations pauvres

concerne, il faut le reconnaître, avant tout des emplois précaires « ubérisés » ; ce ne sont pas les emplois que l'on peut souhaiter pour nos enfants ou pour nos concitoyens.

dont celles-ci ont fait preuve durant la crise, montrant bien leur volonté de contribuer à l'amélioration de la vie quotidienne de nos concitoyens. Enfin, monsieur le ministre, vous ne voyez pas les effets de l'inaction climatique de votre gouvernement, deux fois condamné L'écologie est censée être une priorité du plan de relance, alors que 4,5 milliards d'euros d'autorisations d'engagement prévues au titre du volet écologie n'ont pas été consommés, soit 25 % du budget alloué. Le retard pris par la France dans la mise en oeuvre de sa transition écologique nous conduit à une catastrophe et à une dépendance énergétique mortifère. Les budgets, c'est du fossile à tous les étages, alors que nous devrions redoubler d'efforts et de moyens en faveur du renouvelable et de la sobriété

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, lors de la première lecture de ce texte, je vous expliquais qu'il n'y avait pas de trésor de guerre pour l'État. Aujourd'hui, je vais profiter de cette nouvelle lecture pour nuancer vos affirmations quant à la bonne santé financière des collectivités, lesquelles ne disposent pas davantage d'un trésor de guerre. Si les transferts financiers des collectivités ont été en hausse en 2021, c'est simplement pour compenser ce qui leur a été pris : la première salve de suppression de la part de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) destinée aux régions et le dynamisme de la compensation de cette réforme, la fiscalité transférée pour compenser des mesures de décentralisation ou encore une meilleure consommation des crédits. le dis, monsieur le ministre : il n'y a pas eu de cadeau pour les collectivités. De plus, la fameuse stabilité de la dotation globale de fonctionnement (DGF) est toujours un leurre, puisque ce dispositif n'est toujours pas indexé sur l'inflation. Pis encore, le Gouvernement mélange péréquation verticale et horizontale, par un tour de passe-passe

Les collectivités ont prouvé la solidité de leur budget, mais l'embellie financière de 2021 n'est pas un rebond naturel suivant la crise, les situations sont très variées et de nombreuses recettes ne sont pas revenues à leur niveau passé. À titre d'exemple, la taxe de séjour enregistre une baisse de 24 % entre 2019 et 2021

Les problèmes structurels demeurent, ils se sont aggravés sous le premier mandat d'Emmanuel Macron et perdureront. Le financement des compétences et les compensations d'impôts supprimés sont insuffisants, comme la compensation aux départements de la revalorisation du RSA, votée au gré de l'absence de majorité du Gouvernement à l'Assemblée. Celle-ci est, certes, une avancée, mais représente une goutte d'eau au regard du reste à charge accumulé au fil des années. Les dotations viennent de moins en moins abonder directement les budgets locaux, et sont remplacées par des dispositifs de contractualisation et d'appels à projets préorientés selon les priorités gouvernementales. En plus d'entraîner l'érosion de l'autonomie fiscale des collectivités,

que la baisse de l'offre de service public ou la hausse des impôts et des tarifs. L'État continue d'en demander toujours plus avec moins, nous le voyons aujourd'hui avec la revalorisation du point d'indice, qui n'est toujours pas compensée. Le Gouvernement prend des décisions sans les assumer financièrement, il se déresponsabilise sur le dos des élus locaux, qui payent l'addition. À en croire la communication gouvernementale,

en déficit de trésorerie, par exemple pour financer le fonds de solidarité. En outre, certains des dispositifs ont été payés à cheval sur deux années, comme la prime

Concernant les délais de dépôt du texte évoqués par le rapporteur général et par Hervé Maurey, ainsi que cela a été expliqué en première lecture, ce texte a été déposé lors du premier conseil des ministres suivant les législatives, comme cela avait été le cas en 2007,

en outre, nous souhaitions prendre en compte les derniers chiffres de l'Insee avant de vous présenter ce texte. Il est évidemment préférable que les délais soient un peu plus larges, c'est ce qui se produira en année normale, en dehors des élections législatives.

le cas, par exemple, de la suppression de la taxe d'habitation et des 5 milliards d'euros de baisse de l'impôt sur le revenu qui ont fait suite au grand débat national.

... Laissons donc le Printemps de l'évaluation au printemps et l'automne budgétaire à l'automne ! Je veux vous rassurer, mesdames, messieurs les sénateurs, grâce à l'accord que les deux chambres ont trouvé autour d'une commission le Printemps de l'évaluation est désormais inscrit dans la loi organique qui entrera en vigueur au mois de septembre prochain. Vous aurez ainsi l'occasion de débattre chaque année avec chacun des ministres de l'exécution des budgets de l'année précédente et de la bonne conduite des politiques publiques associées.

le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Les salariés résidant à 30 kilomètres ou plus de leur lieu de travail, ne bénéficiant pas de solution alternative à l'usage de la voiture individuelle et percevant jusqu'à deux SMIC,

mais aussi à celles et ceux qui traversent la France avec leur véhicule pour aller, par exemple, vers l'Espagne ou l'Italie, et qui bénéficieront de la même manière de cet accompagnement financier payé par le contribuable français.

Si nous subventionnons tous les usagers de la même manière, nous allons aggraver notre balance commerciale, singulièrement au mois d'août, lorsque les habitants du nord de l'Europe, transitant par la France pour

le prix de l'essence pour tout le monde, y compris pour ceux qui n'en ont pas besoin, y compris pour ceux qui ont les moyens de supporter cette hausse du prix de l'essence, y compris pour ceux qui se déplacent par convenance personnelle.

En effet, les aides à domicile utilisent leur véhicule personnel afin de se rendre chez les personnes âgées en perte d'autonomie, les personnes en situation de handicap ou les familles en difficulté. parcourent en moyenne, en zone rurale, entre 300 et 400 kilomètres par semaine pour se rendre chez les personnes âgées en perte d'autonomie. L'impact financier de la hausse des prix des carburants est considérable pour elles, dont les salaires sont proches du SMIC. Leur indemnité kilométrique, bien que revalorisée, ne

actuellement le carburant le moins cher disponible à la pompe. Bien qu'il entraîne une consommation supérieure, il est deux fois moins cher que le gazole, le sans plomb 95

M. Guillaume Gontard. Les hypermarchés représentent un modèle aujourd'hui dépassé. Cette révolution du siècle dernier est le symbole des dérèglements de notre temps : surconsommation, étalement urbain, abandon des centres-villes, surutilisation de la voiture,

Il est temps d'en finir avec cette fuite en avant, qui, en plus de bétonner nos terres, tue nos centres-villes, les vide de leurs commerçants et de leurs habitants. Ce modèle entraîne également des dépenses supplémentaires pour les collectivités

Une taxe de même nature a été créée en Île-de-France pour les surfaces de stationnement des hypermarchés et centres commerciaux offrant plus de 2 500 mètres carrés de surface de vente. Cet amendement vise à étendre cette taxe à l'ensemble du territoire afin de participer à la lutte contre l'artificialisation des terres, comme le préconise la Convention citoyenne pour le climat au travers de l'objectif « zéro artificialisation nette

M. Guillaume Gontard. Le régime fiscal applicable aux activités de navigation maritime et au transport de marchandises sur ces voies questionne la pertinence de la politique environnementale française. Responsable d'une pollution dont l'impact environnemental est supérieur à celui de l'automobile, le transport maritime demeure toutefois bénéficiaire d'une exonération de taxe sur les carburants. Alors que l'acheminement de marchandises se fait essentiellement au moyen du fret maritime, les émissions d'oxyde de soufre générées par ce dernier et leurs lourdes conséquences sanitaires et écologiques ne peuvent que contraster avec la faiblesse des réglementations sur les carburants. Afin de rétablir une cohérence dans le traitement de l'urgence environnementale par la France, il est proposé par cet amendement que le fret maritime participe à hauteur de son impact sur les écosystèmes à l'effort fiscal français en faveur de la transition écologique. En ce sens, il est estimé nécessaire que ce secteur soit concerné par les prélèvements de taxe sur les carburants. Alors que les amateurs français, au premier rang desquels CMA CGM, réalisent des profits records- 18 milliards de dollars pour CMA CGM en 2021 -, le maintien de cette exonération paraît d'autant plus aberrant.

ils souhaitent retirer de l'assiette de la TVA des consommations de la fourniture d'eau, de gaz, d'électricité et des carburants les impôts et taxes énergétiques, et ainsi en finir avec la double taxation sur les dépenses d'énergie. Voilà une mesure très simple en faveur

en sortant de l'assiette de TVA la TFCE, la TCA et la TICGN. Cosigné par vingt-neuf de mes collègues de tous bords politiques, cet amendement aura le mérite de clarifier les choses. Je précise, enfin, que j'aurais pu présenter le même amendement

je rappelle que la suppression de la TVA sur les impôts et taxes est contraire au droit européen. Aux termes de l'article 78 de la directive TVA de 2006

! C'est un vrai problème que je vous invite à régler, monsieur le ministre, « quoi qu'il en coûte

devront être fixées dans le cadre du contrat de relance et de transition écologique conclu entre l'État et la collectivité ou le groupement concernés. La région pourrait être cocontractante des contrats avec les collectivités locales de son territoire. Cet amendement régulièrement adopté- et à raison -par notre Haute Assemblée pourrait apporter des subsides concrets à nos collectivités, qui sont toutes en recherche de moyens pour faire face aux investissements qu'impliquent le changement et l'adaptation climatiques. Les collectivités ont un rôle essentiel à jouer dans la planification écologique. Toutes les instances environnementales et tous les experts de notre pays le soulignent : l'action publique locale est l'outil principal du changement. La mesure proposée permet de répondre aux besoins chroniques d'ingénierie territoriale pour atteindre nos objectifs climatiques. Je vous invite donc, mes chers collègues, à renouveler le vote que vous avez déjà émis à de nombreuses reprises.

qui permettra enfin de mettre en oeuvre de manière cohérente les grandes politiques dont nous avons besoin, comme les politiques de rénovation thermique des logements, extraordinairement absentes des deux derniers textes de loi que

entende ce que dit le Président de la République et mette en oeuvre cette contribution climat pour les territoires absolument essentielle à la transition écologique en France

Le plan de relance est une formidable opportunité à la fois pour atteindre nos objectifs climatiques et pour créer de l'activité économique locale ainsi que de l'emploi. Cette mesure s'inscrirait ainsi dans la lignée des orientations annoncées par le Gouvernement en créant

kilomètres de réseaux de chaleur. Les projets en matière de chaleur renouvelable se multiplient, mais la trajectoire actuelle n'est pas suffisamment soutenue pour atteindre les objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. La chaleur représente près de 50 % des besoins énergétiques de la France. Elle est pourtant aujourd'hui massivement produite par des énergies fossiles importées et émettrices de gaz à effet de serre. Afin de se passer rapidement de ces importations dans le contexte du conflit russo-ukrainien et d'atteindre nos objectifs climatiques,

Kern, pour présenter l'amendement n° 53 rectifié. Cet amendement vise à instaurer une écocontribution sur les produits mis sur le marché qui n'entrent dans aucune filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) ou de récupération, réaffectée au financement du service public de gestion des déchets.

conçus à partir de résine vierge. Le Sénat a su en son temps prendre en compte la lutte contre les déchets plastiques, dont nous connaissons les impacts environnementaux néfastes. Rappelons que les metteurs sur le marché visés ici ne contribuent pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché des biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais

en créant une écocontribution qui pourrait utilement inciter à l'utilisation de matières recyclables dans la production même des biens, tout en créant une prise de conscience de la part d'industriels du traitement pour ces futurs déchets. Chacun sait que le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas. Il est donc anormal que cette prise en charge revienne, au bout de compte, aux collectivités locales. Ainsi, pour tous les produits plastiques non couverts par une filière REP, nous demandons la mise en place de cette écocontribution susceptible de permettre de créer une nouvelle recette de la filière REP globale, pour tous les déchets plastiques. Changer notre production est un élément majeur pour une future planification écologique efficace, conforme à notre lutte contre la pollution plastique.

pour nous tous, citoyennes et citoyens, car cette gabegie s'apparente à une certaine forme de gaspillage. Il est temps, enfin, d'aller vers l'économie circulaire et vers une réelle écoconception comme préalable indispensable

Le mécanisme du plafond mordant vise la ponction par l'État des recettes des agences de l'eau au-delà du montant maximum de prélèvement des redevances. Ce principe remet en cause celui de « l'eau paie l'eau » et permet à l'État d'opérer une ponction sur les agences de l'eau. Alors que, dans le cadre du onzième programme des agences de l'eau, celles-ci voient leur champ d'action étendu notamment à la lutte contre le changement climatique, l'institution d'un plafond mordant induira nécessairement la diminution et l'arrêt de certaines aides, pourtant toujours nécessaires pour les territoires. Cet amendement, qui a été travaillé avec l'association Amorce, vise donc à rehausser le plafond mordant pour les agences de l'eau à un niveau correspondant aux moyens annuels dont elles disposaient pour la période 2013-2018, afin d'éviter le report ou la suppression de dispositifs d'aides qui sont nécessaires à la bonne gestion de l'eau dans les territoires. Le maintien du plafond garantit toutefois l'absence de prélèvement supplémentaire. Les agences de l'eau contribueraient ainsi à l'effort budgétaire en intervenant sur des domaines élargis, comme cela a été acté pour le onzième programme, sans disposer de nouveaux moyens.

les produits énergétiques (TICPE) rurale en minorant, à hauteur de 5 %, les tarifs de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que le gaz et le charbon dans les communes situées dans des départements de faible densité de moins de 35 habitants au kilomètre carré et dépourvues de réseau de transport public à l'année.

représenter jusqu'à 5 % du budget des femmes, et ce alors qu'elles sont surreprésentées parmi les faibles revenus et davantage touchées par la précarité et les temps partiels contraints. Alléger cette dépense dans le cadre d'un projet de loi sur le pouvoir d'achat, dans un contexte de tensions inflationnistes, serait donc une mesure spécifique bienvenue. La précarité menstruelle est un enjeu majeur de santé publique,

pratiqués par les industriels du secteur pour que la mesure bénéficie effectivement au pouvoir d'achat des femmes et pour éviter certaines dérives constatées lors de l'abaissement de 20 % à 5,5 % du taux de TVA sur les protections périodiques.

Depuis, la situation a évolué et encore plus de femmes sont dans des situations d'urgence sociale. Ce coup de pouce pour leurs charges contraintes d'hygiène- car il s'agit bien de charges contraintes, au même titre que le loyer et la voiture ! -n'est pas à négliger si l'on veut prendre au sérieux la lutte

estime que 2,6 millions de personnes âgées de plus de 65 ans en souffrent, qu'elles soient hébergées à domicile ou en Ehpad. Pour des raisons de santé publique, il est impératif que ces protections aient un prix abordable. En raison de son coût budgétaire important, l'accès à ces produits est en effet dans les maisons de retraite, comme on a pu le constater. Je tiens d'ailleurs à rappeler que la loi de finances pour 2016 avait étendu le taux de la TVA à 5,5 % aux tampons et aux serviettes périodiques. Il semble juste de l'étendre aux protections hygiéniques pour personnes âgées.

effectuées par les entreprises de moins de 250 personnes et les associations relevant de l'économie sociale et solidaire. L'objectif est de créer un écosystème favorable au développement d'une consommation sobre, ce qui est également, je crois le savoir, le souhait du Gouvernement. Quel est l'avis

en abaissant le taux de TVA à 5,5 %. Nous savons que les transports représentent 31 % des émissions françaises de gaz à effet de serre, premier secteur en termes d'émissions. Une évolution en profondeur de nos modes de déplacements est donc essentielle un report vers des modes de transport décarbonés, peu polluants et générateurs d'externalités positives. L'adoption de cet amendement permettrait de consacrer à nouveau les transports publics du quotidien au rang de service public de première nécessité, comme c'était le cas jusqu'au 1 janvier 2012, avant que la TVA applicable ne soit augmentée à 7 %, puis à 10 % en 2014.

de lutter contre la surconsommation ostentatoire, dont les effets climatiques sont néfastes. L'explosion du patrimoine des milliardaires n'accroît pas seulement les inégalités sociales : elle est néfaste pour le climat, et même pour le climat social. En effet, selon le rapport sur les inégalités mondiales, l'empreinte carbone des 1 % les plus aisés est quinze fois plus élevée que celle des cinq premiers déciles. Tout le monde peut se moquer de l'accord de Paris que nous avons signé et du devenir du climat. Pour notre part, nous proposons, avec cet amendement, amendement, de taxer plus fortement et d'inciter à la sobriété.

le taux de TVA à 2,1 % également pour les produits alimentaires issus des circuits courts. Je ne développerai pas plus avant mon

Renforcés dans nos convictions par les travaux de la Convention citoyenne, nous reformulons la proposition d'une TVA à 2,1 % pour le vrac alimentaire et à 10 % pour le vrac non alimentaire. Cette filière, qui répond à une réelle demande des consommateurs et consommatrices, peine à se déployer pleinement. Afin de renforcer son attractivité et de s'assurer qu'elle participe au renforcement du pouvoir d'achat des consommatrices et consommateurs, nous proposons, dans le cadre de la loi de finances, d'agir sur le taux de TVA applicable aux produits non emballés. Ainsi, nous proposons d'appliquer le taux de TVA super réduit de 2,1 % aux produits alimentaires vendus en vrac, et le taux de 5,5 % pour le reste. Nous proposons également de fixer un taux de TVA des produits non alimentaires à 10 % au lieu de 20 %. Il s'agit d'un exemple concret permettant de conjuguer exigences sociales et écologiques, en rendant financièrement accessible ce qui est écologiquement responsable. Il faudra ensuite, comme cela vient d'être rappelé, que le Gouvernement porte cette exigence auprès des instances européennes afin de les rendre effectives. Quel

les coupures d'eau sont récurrentes

d'inciter leurs propriétaires à les occuper, à les vendre ou à les louer. Les taux de la taxe annuelle sur les logements vacants étant notoirement insuffisants, nous proposons de les augmenter, afin d'obtenir des résultats plus probants en matière d'occupation des logements vacants.

revenues à leur niveau de 2019. Évidemment, il n'y a pas de trésor de guerre dans les collectivités territoriales. Eh non ! Cela se saurait ! Les élus locaux demandent donc de la visibilité pour pouvoir continuer de faire vivre les services publics locaux et d'être moteurs de l'investissement public, ce qui est très important.

ouverte et constructive, en nous efforçant de cibler les aides sur les collectivités qui en ont le plus besoin.

favorable.

Le président du Sivom Val de Banquière, dans les Alpes-Maritimes, et le maire de la commune de La Trinité ont alors introduit une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel,

mais il y en a bien d'autres dans d'autres départements -, qui ont ainsi pu continuer à assurer leur mission de proximité sans avoir à grever leur budget.

du point d'indice des fonctionnaires et à l'inflation qui touche de nombreux produits énergétiques ou alimentaires. Les nombreux amendements qui vont être présentés témoignent, s'il en était besoin, de notre volonté commune de soutenir les collectivités. Nous étions en droit de nous étonner que le Gouvernement,

Au regard des contraintes que l'inflation fait peser sur le maintien de services publics comme les cantines scolaires, par exemple, je propose là aussi d'élargir l'assiette aux dépenses de produits alimentaires avec un taux de compensation de 70 %. Mon amendement tend également à porter de 50 % à 70 % la compensation de la hausse des produits énergétiques. Les communes seraient ainsi compensées au travers de l'article 4 et les départements au travers Pour compléter le dispositif, je présenterai l'amendement n° 544 visant à soutenir les régions en compensant la revalorisation de 4 % des rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle. L'ensemble de ces dispositifs représente un soutien financier total d'environ 750 millions d'euros. Le paquet de mesures, si j'ose dire, proposé par la commission est plus complet que le texte initial dans la mesure où il s'adresse à toutes les collectivités locales.

les collèges, les infrastructures routières, le développement des pratiques culturelles et sportives ... Sans compensation, il leur faudrait renoncer à des investissements cruciaux, ou

Le sous-amendement vise, comme certains sénateurs le souhaitaient, à mieux cibler l'aide apportée aux régions, dont les recettes de TVA ont augmenté de plus de 2 milliards d'euros.

aux collectivités bénéficiaires du Fonds de solidarité, au titre de la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle. Il s'agit, en l'occurrence, comme vous l'avez rappelé, des régions d'outre-mer et de la Corse.

accès aux compensations. La

En quoi le sous-amendement du Gouvernement le gêne-t-il ? Son amendement se suffit-il en lui-même ? Pourrait-il se passer du sous-amendement du Gouvernement ?

pardonnerez de penser que l'article 4, arraché de justesse à l'Assemblée nationale et évalué à 180 millions d'euros, ne fait pas la maille. À côté de solutions pérennes, comme le rétablissement du bénéfice des tarifs réglementés de vente de l'énergie, nous proposons une solution d'urgence, pour 2022, avec une dotation énergie de soutien aux collectivités pour faire face au surcoût.

à titre exceptionnel, de l'ordre de 600 000 euros, pour appuyer la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui doit faire face à une hausse substantielle de sa facture énergétique, de l'ordre de 60 Ces dépenses énergétiques supplémentaires et imprévues sont de nature à affecter le budget de la collectivité, en particulier son volet investissement, lequel doit être préservé au niveau actuel, afin de maintenir l'attrait de la collectivité dans une ère post-covid. L'auteur de cet amendement souhaite en particulier attirer l'attention du Gouvernement sur la spécificité de l'archipel. L'insularité conduit à des dépenses énergétiques particulières, puisque la collectivité dispose notamment de deux navires de type ferry, indispensables pour le territoire. En conséquence, les dépenses liées au fuel ont considérablement augmenté. Il est donc demandé de créer un prélèvement sur recettes « bouclier énergétique Saint-Pierre-et-Miquelon », afin d'apporter une aide temporaire, mais décisive, à cette collectivité. Quel est l'avis de

en métropole et dans la plupart des départements d'outre-mer, voire davantage dans certains départements d'outre-mer. À Saint-Pierre-et-Miquelon, les circuits d'approvisionnement, qui sont liés à l'Amérique du Nord, font que les prix énergétiques auraient beaucoup moins augmenté que dans le reste du territoire national.

choses, quand l'État décide en lieu et place des collectivités locales, est d'assumer lui-même le coût de ses décisions. C'est une question de méthode. La revalorisation

fonction publique territoriale va devoir assumer une part importante de la réévaluation des traitements des agents publics. Si je tiens à souligner que ce rehaussement du point d'indice constitue une mesure minimale après des années de gel, n'en est pas moins difficile à assumer pour des collectivités territoriales dont les finances ont été amoindries d'année en année et qui font face au choc énergétique.

ma collègue Maryse Carrère. La revalorisation du point d'indice de la fonction publique décidée par le Gouvernement, pour légitime qu'elle soit, a des conséquences financières préjudiciables pour les collectivités locales, plus particulièrement les communes et leurs groupements. La décision de revaloriser de 3,5 % le point d'indice depuis le 1 juillet dernier représente un surcoût pour les collectivités locales estimé à 2,27 milliards d'euros en année pleine,

découle d'une décision gouvernementale, dont la responsabilité financière est reportée sur les collectivités, tandis que l'autre est la conséquence de l'inflation et de l'absence de mesures protectrices suffisantes pour limiter les hausses pour les collectivités. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de traiter ces deux aspects par le biais d'amendements distincts.

d'autofinancement. En effet, ce critère apparaît comme un meilleur indicateur de santé financière des collectivités. La capacité d'autofinancement, lorsqu'elle est positive, est égale à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. Elle permet de rembourser les annuités de dette et de financer les dépenses d'équipement propres et les subventions d'équipement. Cet amendement prévoit également une amélioration rédactionnelle par la suppression du mot « principalement », qui n'a pas de portée juridique.

à 20 %. Cela permettra de rendre potentiellement éligibles à la dotation de soutien près de 50 % des communes et de leurs groupements, contre environ 20 % avec l'article 4 actuel. Par ailleurs, la rédaction retenue prévoit une compensation à hauteur de 50 % de la hausse des dépenses liées, d'une part, à la revalorisation du point d'indice, d'autre part, à l'inflation des produits énergétiques. Nous proposons de porter ce pourcentage de 50 % à 70 %.

pour le bloc communal, est évalué à plus de 600 millions d'euros. J'ai dit être équitable et magnanime, mais il faut aussi être raisonnable, tout en

Je me réjouis que notre groupe ait pris part au compromis trouvé cet après-midi par le Gouvernement et le rapporteur général. Il était essentiel d'apporter un soutien fort de l'État aux collectivités du bloc communal, les plus touchées par la revalorisation du point d'indice de la fonction publique et par l'inflation des prix de l'énergie.

Monsieur le ministre,

Par cet amendement, nous proposons la création d'une dotation de soutien aux collectivités qui font face à une augmentation de leurs dépenses de restauration collective due à l'inflation. Selon Restau'co, qui fédère la restauration collective en gestion directe, sans action de l'État, les budgets des cantines scolaires pour 2022 auront été consommés à la mi-septembre, juste après la rentrée. En effet, du fait de la forte inflation, qui vient de passer la barre des 6 %, le coût moyen des plateaux-repas dans les cantines a augmenté de 5 % à 10 % ; il arrive même que l'augmentation atteigne 15 %, selon l'association des gestionnaires de cantines scolaires.

Cet amendement vise donc à compenser une partie des investissements réalisés par les régions pour le développement des infrastructures de transports publics. La mise en commun des modes de transport et la promotion des mobilités partagées permettront d'atténuer les effets de l'inflation, qui touche en particulier les prix de l'essence. Il est proposé, à cette fin, d'instituer une dotation abondée à hauteur de 500 millions d'euros.

mais ce n'est pas comme si l'État avait décidé tout seul, dans son coin, du périmètre du remboursement.

à agir de nos collectivités. Instaurer la contemporanéité du FCTVA constituerait un signal positif envoyé aux élus locaux, à l'heure où des investissements massifs sont nécessaires.

pour les autres élus locaux, notamment la prise en charge des frais de garde, un droit à la formation et à un bilan de compétence à la fin de leur mandat ou encore l'éligibilité à une allocation différentielle de fin de mandat. Cette démarche vise

à financer des mesures améliorant le statut des élus locaux, notamment la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints, les autorisations d'absence et les frais de formation des élus. Cette dotation est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants, sous condition

DPEL. Pour atteindre cet objectif, tout en conservant les attributions individuelles à leur niveau actuel, nous proposons de relever le volume total de la dotation à 114,7 millions d'euros, contre 101 millions d'euros actuellement. La parole